afin de respecter les règles sanitaires, je vous rappelle que le port du masque est obligatoire dans l'enceinte du palais et qu'il vous est demandé de laisser un siège vide entre deux sièges occupés. L'hémicycle fait bien sûr l'objet d'un nettoyage et d'une désinfection en profondeur chaque semaine, que les micros sont chaque fois désinfectés. Chacun veillera au respect des distances de sécurité. Les sorties de la salle des séances devront exclusivement s'effectuer par les portes situées au pourtour de l'hémicycle, à l'exception de celles des membres du Gouvernement,

À l'heure où le Président de la République s'apprête vraisemblablement à durcir les mesures sanitaires pour faire face à la deuxième vague de la covid-19, je voudrais surtout vous parler de leur impact social. C'est un véritable drame que vivent des centaines de milliers de familles françaises : 715 000 emplois ont été détruits au premier semestre, et, d'ici à la fin de l'année, nous serons vraisemblablement non loin L'approche que nous avons eue de la pandémie fera sombrer de très nombreux ménages déjà précaires dans l'extrême pauvreté et les classes moyennes dans la précarité. Le pays est inquiet, vous le savez. Votre tâche n'est pas facile, mais c'est vous qui êtes aux responsabilités. C'est bien pourquoi il ne faut pas seulement recalibrer le volet sanitaire ; nous vous invitons aussi à recalibrer le soutien à l'économie. La deuxième vague de la pandémie impose d'accélérer en parallèle le plan de relance. Dès le mois de juillet le Sénat vous avait alerté sur la nécessité d'agir tout de suite, comme l'ont fait nos voisins allemands et anglais, mais le plan de relance n'a cessé d'être différé. Lors de l'examen du projet de loi de finances rectificative 2, il avait été annoncé que ces mesures seraient mises en oeuvre dès le PLFR 3. À l'occasion de ce PLFR 3, il nous a été annoncé qu'elles le seraient dans un PLFR 4. Or ce PLFR 4 n'est jamais arrivé. Le plan de relance est finalement porté par le budget pour 2021, donc concrètement différé au début de l'année prochaine. Cela va nous conduire à dégainer avec plusieurs mois de retard ... Nos concitoyens ne peuvent pas attendre : de nombreux commerces, de nombreux artisans, des TPE, des PME ne tiendront pas encore trois mois. Des secteurs entiers se trouvent dans une extrême difficulté. Dans ces conditions, monsieur le Premier ministre, allez-vous accélérer la mise en oeuvre du plan de relance, et si oui, comment ? La parole est à M. le Premier ministre. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, vous me permettrez tout d'abord d'adresser, au nom du Gouvernement, mes plus sincères félicitations aux nouvelles sénatrices et aux nouveaux sénateurs qui ont rejoint, à la faveur du dernier scrutin, le Palais du Luxembourg. Je voudrais également, monsieur le président, vous adresser mes félicitations personnelles pour votre brillante réélection à la tête de la Haute Assemblée. Monsieur Monsieur le président Hervé Marseille, vous l'avez dit, la situation de notre pays est extrêmement difficile.

forte. Vous l'avez également souligné, elle va conduire le Gouvernement, dans la continuité des dispositions qu'il a prises, à adopter des mesures complémentaires pour faire face à cette situation. Vous avez raison, le Président de la République aura l'occasion d'y revenir dès ce soir.

à engager des moyens- 470 milliards d'euros, très précisément -dès le début de la crise, pour faire face à ses conséquences économiques et sociales.

Je me permets d'indiquer à la Haute Assemblée que les secteurs les plus touchés, en particulier- pour faire le lien direct avec les mesures à caractère sanitaire -tous les secteurs professionnels qui sont concernés par la mise en oeuvre des mesures administratives qu'appelle la présente situation, font l'objet de mesures extrêmement précises

économique, je précise à la Haute Assemblée- c'est un élément essentiel de notre stratégie -que nous prenons et allons continuer à prendre les mesures de protection sanitaire que la situation exige.

prochain, à l'occasion de la journée internationale de lutte contre la misère, après la concertation, j'annoncerai un certain nombre de mesures que les circonstances actuelles exigent. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs,

rassemblement et sens des responsabilités, le Gouvernement tout entier, derrière le Président de la République, est mobilisé et déterminé. La parole et de la santé. Monsieur le ministre, en cette période de rebond de pandémie de la covid-19, notre système de santé est de nouveau sous tension. Tous les voyants sont au rouge. Vous assurez maîtriser la situation. Le Président de la République va faire des annonces ce soir, orientées visiblement vers de nouvelles restrictions de libertés, ce n'est pas la solution. Vous n'avez pas tiré les leçons de la première vague, et de nouveau les hôpitaux sont saturés. Les personnels soignants crient leur inquiétude et leur colère. Ils sont épuisés, démunis, sous-payés, avec des directions de plus en plus autoritaires, et on leur demande de faire face de nouveau. Cette fois, la pandémie se répand partout partout sur le territoire ; cette fois, il n'y aura pas de renforts de personnels pour aller au secours de telle ou telle région débordée. Et l'hôpital n'a toujours pas les moyens nécessaires pour faire face de nouveau à un manque insupportable de lits et de personnels. Quant à la médecine de ville, elle est aussi en difficulté. Aussi, ma question est simple, monsieur le ministre : que dites-vous aux personnels hospitaliers qui seront dans la rue demain pour dire que le Ségur ne fait pas le compte ? Que dites-vous à toutes celles et à tous ceux qui démissionnent, des chefs de service- je pense notamment au docteur Maurice Raphaël, chef des urgences de l'hôpital Bicêtre depuis dix ans -, jusqu'aux infirmières et aux aides-soignantes

Madame la sénatrice, à entendre le début de votre question, je me suis presque demandé si l'on parlait bien d'une épidémie causée par un virus circulant en France, en Europe et dans le reste du monde,

Madame la sénatrice, dans quelques jours, dans quelques semaines, vous voterez- je l'espère -un projet de loi de financement de la sécurité sociale qui porte en lui-même le renouveau de l'hôpital public : création de 4 000 lits- alors que, jusqu'à présent, on en fermait des milliers tous les ans embauche de 15 000 soignants à l'hôpital- alors que cela fait des années que la masse salariale n'était plus adaptée à la charge de travail -, sortie de la tarification à l'activité pour aller vers une dotation populationnelle, changements des règles de gouvernance internes aux établissements de santé, pour permettre une meilleure représentativité des professionnels de santé en leur sein, enfin-

progressistes et indépendants. Ma question s'adresse à M. le ministre de l'Europe et des affaires étrangères. Monsieur le ministre, il n'est pas besoin de rappeler ici la longue histoire d'amitié qui unit la France et l'Arménie et l'affection que nous portons à nos amis arméniens. De nombreuses villes de mon département, la Drôme, mais aussi du Rhône, de l'Isère et des régions parisienne et marseillaise ont tissé des liens étroits avec le Haut-Karabakh, en raison des liens de fraternité entre Français et Arméniens. Une belle illustration en est la signature d'une charte d'amitié entre le département de la Drôme et le Haut-Karabakh en 2015. Le 27 septembre 2020, nous avons assisté impuissants à l'entrée en conflit de l'Azerbaïdjan contre les Arméniens du Haut-Karabakh. Cette offensive militaire est venue brutalement raviver le « conflit gelé » autour de ce territoire, qui bénéficiait, depuis l'accord de cessez-le-feu de 1994, d'une relative stabilité, certes marquée par des épisodes de tension. Aujourd'hui, avec la nouvelle violation de ce cessez-le-feu, notre inquiétude est grande. Nous constatons des affrontements d'une extraordinaire violence, qui se développent non seulement le long de la ligne de front, mais aussi dans nos villes amies : Stepanakert- amie avec la ville de Valence -, Chouchi, Martuni. Les premières victimes en sont les populations civiles, des familles arméniennes que nous connaissons bien. Je sais, monsieur le ministre, que, dans le cadre du groupe de Minsk, vous ne ménagez pas vos efforts pour résoudre ce conflit et pour aboutir à une solution garantissant la paix et la sécurité des populations civiles. Toutefois, notre préoccupation est vive quand nous voyons que le cessez-le-feu humanitaire négocié samedi dernier peine, lui aussi, à être respecté. Dans de nombreuses villes de France, et hier soir à Paris, nous avons affirmé, nombreux, notre entier soutien au peuple arménien et karabahiote, ainsi que notre indéfectible amitié. Monsieur le ministre, que peut faire la France pour arrêter cette offensive de l'Azerbaïdjan, qui est meurtrière pour les populations civiles d'Artsakh ? Je vous remercie par avance de votre réponse.

Une urgence, parce que l'escalade qui se poursuit entraîne de nouvelles victimes, particulièrement des victimes civiles. Cette situation suscite une émotion légitime, en particulier en France, du fait de la proximité des liens humains, des liens culturels, des liens historiques qui nous lient à l'Arménie. Vous avez fait part de cette émotion, que je comprends et que je partage. Cette émotion, elle justifie que nous accentuions encore nos efforts pour faire accepter l'arrangement qui est intervenu samedi à Moscou, en notre présence, pour aboutir à un cessez-le-feu. Il y a urgence, parce que les ingérences étrangères, en particulier celle de la Turquie, alimentent cette escalade. Elles ne sont pas acceptables. Il y a aussi un devoir, celui du mandat que nous a confié l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, l'OSCE, dans le cadre du groupe de Minsk, que vous avez cité et que nous coprésidons avec la Russie et les États-Unis. Nos efforts se poursuivent en permanence, y compris, monsieur le sénateur, en ce moment même à Erevan et à Bakou.

Et à ceux qui souhaitent voir la France y renoncer, je dis que l'amitié qui nous lie à l'Arménie, au peuple arménien, serait mal servie si nous renoncions à ce rôle d'équilibre, perdre notre impartialité, ce serait aussi laisser la porte ouverte à un rôle plus direct de la Turquie dans le règlement de la crise. Or il n'est pas possible qu'un pays puisse être à la fois protagoniste d'un conflit et partie prenante de son règlement.

Ce constat, nous le faisons collectivement depuis de nombreux mois, et il vient malheureusement d'être confirmé par ce chiffre dramatique : la crise sanitaire, mes chers collègues, a fait basculer 1 million de Français dans la pauvreté. Ils rejoignent les 9 millions de nos concitoyens qui vivaient déjà sous le seuil de pauvreté. Dans le même temps, un rapport de France Stratégie nous informe que la suppression de l'impôt sur la fortune et l'instauration de la au début du quinquennat ont eu pour effet de faire fortement augmenter les revenus des 0,1 % des Français les plus aisés, tandis que la distribution de dividendes, de plus en plus ciblée, a explosé. Cette concentration du capital n'est pas acceptable. Elle l'est encore moins quand tant de Français sont dans la souffrance. Votre politique aggrave les inégalités sociales et territoriales. Vous auriez dû agir ; il est trop tard. Je vous demande donc de réagir. Ainsi, je fais un rêve : celui d'un gouvernement capable de revenir sur ses erreurs, de supprimer son bouclier fiscal, devenu un tremplin fiscal, et de penser à de nouvelles ressources liées à la taxation du capital celui d'un gouvernement qui ouvre le revenu minimum aux jeunes pour les empêcher de sombrer ; celui d'un gouvernement qui abroge sa réforme de l'aide personnalisée au logement, l'APL, qui revalorise le point d'indice pour les agents de la fonction publique et qui donne un coup de pouce au SMIC. En somme, je fais le rêve d'un gouvernement qui lutte enfin contre les inégalités, qui dégrippe l'ascenseur social et qui empêche de nouvelles catégories de la population de tomber dans la précarité. Monsieur le Premier ministre, la réalité est là, sous vos yeux, sous nos yeux, tragique. Allez-vous la prendre en compte et enfin changer de cap ?

grâce à une baisse des impôts, la croissance en France était l'une des meilleures de l'Union européenne, le niveau de chômage était également l'un des plus satisfaisants, tandis que les investissements étrangers n'avaient jamais été aussi nombreux depuis dix ans. Bref, cher président Kanner, des résultats économiques nettement supérieurs à ceux que vous aviez enregistrés à la fin du précédent quinquennat

et des chiffres du chômage et, hélas, de ceux de la pauvreté. Je rappelle au Sénat que notre système de protection sociale

à destination de ces publics. Une aide exceptionnelle de solidarité a été versée le 15 mai dernier à 4,1 millions de foyers en difficulté,

les plus démunis dans la crise. Cette réponse sera à la hauteur, mais elle n'invalide pas notre politique de fond, qui, plutôt que d'installer des gens dans les allocations, vise à les insérer

Monsieur le Premier ministre, votre réponse ne définit pas une politique, c'est un slogan ! J'ai le sentiment que, quand les Français tombent,

obtenu depuis le début de ce quinquennat n'aurait pas été scandaleux. Vous vous y refusez : je tiens à vous dire que les Français sauront vous juger.

Dès le mois de juillet, tout le monde s'accordait à dire que nous allions vivre une nouvelle vague de l'épidémie. Ça y est, nous y sommes ! La métropole de Montpellier, dans mon département, vient de rejoindre la liste des territoires en alerte maximale Covid.

d'un manque de moyens financiers ou de personnel compétent ? Pourquoi ne pas avoir pensé à une stratégie d'urgence ? J'ai conscience que la situation n'est pas facile, mais les Français ne comprennent pas. Il faut leur expliquer simplement. À la crise sanitaire, on répond par des mesures liberticides, mais on ne traite pas la problématique des moyens de l'hôpital public. Pour ma part, je suis pragmatique : quand un tuyau a trop de pression et risque de céder, on ne coupe pas l'eau, Sur le terrain, certains médecins généralistes se plaignent du manque de communication et de cohérence avec les hôpitaux. Ils craignent des retards dans la prise en charge des autres pathologies.

Tout cela provoque une véritable inquiétude face à l'épuisement, voire au burn-out de certains personnels. Quelles mesures allez-vous prendre pour soulager les soignants, qu'ils soient sur le terrain ou dans les établissements ? Vous avez raison de penser à eux, nous y pensons aussi, mais je crains que cela ne suffise

En revanche, nous avons formé du personnel pour qu'il puisse aider en réanimation. Rien qu'en Île-de-France, ces derniers mois, 750 infirmières sont venues en service de réanimation ou en apprentissage par simulation, pour prêter main-forte à leurs collègues si la situation l'exigeait. Hélas, on ne trouve pas

Ma question s'adresse à M. le Premier ministre. Pour faire face à une crise économique, sociale et climatique d'une ampleur sans précédent, l'Union européenne a adopté un plan de relance historique de 750 milliards d'euros. Malheureusement, en contrepartie, le cadre budgétaire 2021-2027 est revu à la baisse. Déshabiller Paul pour habiller Jacques n'a jamais fait une politique ambitieuse ! Pour financer la relance européenne, il faut, au contraire, renforcer les ressources propres de l'Union.

Faire contribuer à l'effort les pollueurs, les multinationales qui se soustraient à l'impôt et la finance débridée, quoi de plus juste ? On se demande vraiment pourquoi rien ne bouge depuis des décennies. Il faut dire que la France, qui a longtemps porté la TTF, n'a jamais été au rendez-vous de son histoire. En 2014, c'est Pierre Moscovici qui torpillait le projet proposé par une Commission de droite, pour défendre le seul intérêt des grandes banques françaises. L'actuel président de la République n'a pas fait mieux. Il a d'abord refusé l'élargissement de la TTF française, avant de plaider pour une TTF européenne, en prenant modèle sur celle du Royaume-Uni- un simple impôt boursier. Depuis lors, rien ou presque, si ce n'est ce projet d'une microtaxe de 0,2 % sur le prix d'achat des actions, qui rapporte seulement 3,5 milliards d'euros par an, soit dix fois moins que le projet de 2013. 2013. Monsieur le Premier ministre, lors du Conseil de demain, le Président de la République va-t-il tout faire pour obtenir des ressources propres ambitieuses, dont la TTF, ou va-t-il se contenter de mots, au détriment de l'intérêt général européen ? La parole est à M. le Premier ministre.

mais que, comme chacun le comprendra, compte tenu de l'objet même de ce prélèvement, c'est le niveau européen qui est le plus approprié.

de la relance des négociations sur la taxe sur les transactions financières européennes, lesquelles négociations avaient effectivement été interrompues sous le précédent quinquennat.

toujours pleine et entière. Il en ira de même sur un autre sujet que vous avez évoqué et qui figure dans les objectifs de transition écologique,

les difficultés rencontrées parce que l'Europe est une union d'États et que l'on ne peut pas décider unilatéralement. Il faut donc encore plus de force de conviction et de volonté, comme en ont eu

beaucoup de travail à faire en la matière, mais, là encore, ne doutez ni de notre détermination ni de la volonté de la France à porter dans le concert européen ce qui relève finalement de l'intérêt de nos concitoyens. La parole

opérant, notamment, des transferts de compétence entre les collectivités territoriales. Les élus locaux ne sont pas près de les oublier : en fait, ils peinent encore à s'en remettre. l'esprit, en particulier, les élus fraîchement arrivés aux responsabilités, en juillet dernier, qui doivent gérer de front l'application des consignes sanitaires et celle des lois votées lors du précédent quinquennat.

le deviendront de plein droit au 1 janvier 2021, sauf à ce qu'un nombre significatif de communes s'y opposent au cours des trois mois précédents. Je vous rassure,

en permettant aux communautés d'agglomération de déléguer, dans un certain délai, tout ou partie de leurs compétences aux communes ou aux syndicats. Or, là encore, ce délai expire au 31 décembre prochain. Ce sont deux exemples d'un même problème : les élus locaux n'ont pas eu de temps à consacrer à ces questions,

de l'Aube et d'ailleurs, de prendre leurs décisions de façon libre et éclairée ? Un report de ces deux échéances vous paraît-il envisageable ? La parole

notamment assoupli et adapté les modalités de transfert en matière d'eau et d'assainissement. Les intercommunalités peuvent désormais déléguer leur compétence aux communes, et cela sans délai : il n'y a pas de date barrière. Je précise, par ailleurs, que les communes peuvent elles-mêmes faire une demande de délégation. Dans cette hypothèse, l'intercommunalité a trois mois pour se prononcer.

sauf si une minorité de blocage a été réunie. Avec la crise sanitaire et le décalage des élections, ce délai a été mécaniquement raccourci, je vous l'accorde. Or je partage l'idée que, pour faire valoir, ou non, son opposition à un transfert, une commune doit disposer de suffisamment de temps pour échanger avec son EPCI.

je vous remercie Ma question s'adresse à M. le Premier ministre et porte sur la Nouvelle-Calédonie. Le 4 octobre dernier, les Calédoniens ont de nouveau rejeté l'indépendance à l'occasion du second référendum ; il va y en avoir un troisième. Le premier effet de ces référendums

aucune perspective n'est ouverte. Il me semble que le Gouvernement confond trop facilement impartialité et indifférence à l'avenir de ce territoire. Il ne s'engage pas. Il ne joue pas son rôle d'arbitre, ne contribue pas, avec les parties calédoniennes, à définir des perspectives allant au-delà de ces référendums à répétition. Avec les accords de Nouméa, nous avons connu une période de plus de vingt ans durant laquelle on pouvait construire. Que peut-on construire aujourd'hui, alors que chacun retient son souffle ? La question que je veux vous poser, monsieur le Premier ministre, est la suivante : le Gouvernement va-t-il enfin s'engager à jouer pleinement son rôle pour fédérer les énergies calédoniennes, afin de définir un avenir qui dépasse l'échéance d'un éventuel prochain référendum inscrit dans la loi organique

tant dans la campagne électorale que dans l'organisation du scrutin. C'était notre première mission dans ce deuxième référendum, et nous y avons veillé scrupuleusement.

Dès cette semaine, à ma demande et en accord avec le Président de la République, le ministre chargé des outre-mer, Sébastien Lecornu, est parti pour le Caillou, où il va rester un certain temps, pour reprendre le fil du dialogue et examiner les voies du développement de la Nouvelle-Calédonie. Ce n'est, vous le savez, qu'à partir d'avril prochain que le Congrès pourra réclamer officiellement l'organisation d'un troisième référendum.

d'organiser les discussions sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Nous le ferons sans tabou, en exposant bien les conséquences réelles

Monsieur le Premier ministre, je ne suis pas convaincu que vous soyez actuellement porteur d'une vision d'avenir pour la Nouvelle-Calédonie qui dépasserait l'échéance d'un éventuel troisième référendum ... Ça, c'est sûr ! Ce butoir que nous avons face à nous n'est en effet pas la fin de l'Histoire, et il faut d'ores et déjà que l'État soit capable, comme le demande avec insistance notre collègue Pierre Frogier, que vous gagneriez à écouter davantage et qui est l'un des signataires des accords de Nouméa, un avenir et d'ouvrir des perspectives. On va le faire ! Vous ne pouvez pas rester simple spectateur à l'abri de la neutralité dont vous devez faire preuve dans le processus électoral. Vous êtes responsable, vous ne pouvez pas rester indifférent. Réunissez à Paris les Calédoniens et donnez-leur des perspectives

et de la relance. Le groupe Veolia, leader mondial des services de gestion de l'eau, des déchets et de l'énergie, s'est lancé dans une opération agressive de rachat de son grand rival français, Suez. Après deux tentatives sans lendemain en 2006 et 2012, le groupe Engie a accepté de vendre à Veolia ses parts de Suez. Cette initiative hostile interroge, d'abord parce que l'argument qui consiste à vanter la création d'un géant mondial est très relatif : réunies, les deux entreprises représenteront moins de 5 % du marché mondial. La France a deux grands groupes sur ce marché ; demain, elle n'en aura plus qu'un. L'opération pourrait s'apparenter davantage au dépeçage d'une entreprise qu'à l'addition de deux groupes. Ensuite, le bénéfice en matière d'emplois d'une telle évolution est difficile à percevoir. Quel sort réservera Veolia aux 30 000 collaborateurs de Suez en France ? Si l'on regarde Alcatel Lucent, Lafarge Holcim ou General Electric Alstom, des promesses ont été faites, mais les synergies annoncées se sont traduites par des plans sociaux. C'est vrai ! Enfin, cette opération va limiter la saine et indispensable concurrence qui existe sur ces marchés au bénéfice des collectivités locales et des citoyens. Veolia et Suez sont deux acteurs importants en concurrence frontale, quoi de plus stimulant ? Ce secteur est connu pour présenter, déjà, des niveaux de concentration élevés. Est-il raisonnable d'aller plus loin ? Est-il raisonnable de faire intervenir un fonds de pension sur un marché où la vision stratégique à long terme est essentielle ?

précédemment évoquées ? Peut-il nous assurer que, contrairement à ce qu'on lit et entend parfois, l'État n'a pas, sur ce dossier, un double langage, hostile au rachat en apparence, mais facilitateur en coulisses ?

Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur Babary, Veolia et Suez sont deux champions français du traitement des déchets et de la gestion de l'eau, présents partout dans le monde. Les Français connaissent bien ces deux entreprises et leur font confiance au quotidien. Nous ne pouvons pas accepter que ces deux champions industriels français se livrent une guerre en plein coeur de l'une des crises économiques les plus graves qu'ait traversées le pays. Nous avions besoin, au contraire, que ces deux industriels prennent le temps de se parler et d'échanger sur un projet qui soit accepté par toutes les parties. Pour être un succès pour Veolia et pour Suez comme pour leurs clients et leurs salariés, cette opération ne devait pas être réalisée en force et dans la précipitation.

alors que les salariés de Suez, notamment plus de 30 000 femmes et hommes employés en France, ont été en première ligne durant la crise pour garantir le bon fonctionnement des services publics essentiels, comme le traitement des déchets ou l'accès à l'eau. La logique industrielle, ensuite, notamment en s'assurant que les acteurs susceptibles de reprendre les activités de Suez en France sont crédibles, robustes et engagés à long terme. Il n'est pas question que cette opération soit le prélude à une perte de souveraineté dans des secteurs sensibles et stratégiques. La préservation d'une offre concurrentielle et de qualité pour remplir les missions essentielles qui relèvent de la compétence l'intérêt patrimonial de l'État, actionnaire d'Engie. Tels sont les critères que Bruno Le Maire a posés d'emblée et qui ont guidé le choix de l'État au conseil d'administration d'Engie. Faute d'accord entre Suez et Veolia, l'État ne pouvait pas valider cette session, qui n'était pas acceptée par l'ensemble des parties prenantes, notamment par les salariés de Suez.

est un camouflet sans précédent sous la V République ! À ce titre, votre immobilisme m'interpelle grandement, car, en temps normal, cet événement aurait dû déclencher un séisme et une réaction immédiate de l'État actionnaire. Je m'interroge : comment l'État peut-il accepter d'être mis en minorité de cette façon sur une question aussi importante ? De ce point de vue, votre attitude dans ce dossier est, pour le moins, très ambiguë : vous semblez avoir agi, si je puis me permettre, à l'insu de votre plein gré non seulement vous n'avez pas fait grand-chose pour empêcher cette OPA, mais, en plus, vous vous êtes empressé de justifier votre impuissance dans la presse. Avec le macronisme, nous vous savions disruptif, mais tout de même Quelle étrange situation : le premier actionnaire d'un groupe, qui en nomme le président, n'est pas capable de se faire entendre ... Nous pourrions presque en sourire, si la situation que votre immobilisme a créée n'était pas si grave 10 000 emplois vont être détruits dans le monde à la suite de ce rachat. À l'heure où la gestion de l'eau et des déchets représente des enjeux capitaux sur les plans économique, social et écologique, comment laisser faire la création d'une entreprise privée, que vous placez, par votre inaction, en position quasi monopolistique, privant ainsi les élus locaux de la possibilité de faire jouer une quelconque concurrence ?

Nous insistons pour que les dirigeants de ces entreprises s'entendent : c'est dans l'intérêt de leur entreprise, des salariés de Suez et des collectivités territoriales, pour lesquelles ces entreprises assurent un service public essentiel. Nous sommes et resterons vigilants sur la suite des événements.

la France subit une vague sans précédent de violences brutales et barbares : un commissariat attaqué à Champigny-sur-Marne, quatre policiers en civil attaqués, hier, en plein jour et à proximité d'une école maternelle, à Montbéliard cette nuit, à Savigny-sur-Orge, dans mon département du Val-d'Oise, deux policiers se sont fait tirer dessus par des individus qui, selon des avocats, les auraient « pris pour des gitans déguisés en flics » ... Admirable et tragique illustration du fameux vivre-ensemble Pendant ce temps, au lieu d'agir, vos ministres s'empêtrent dans des querelles aussi irréelles que celles des théologiens de Byzance quand les Ottomans étaient aux portes de la ville : le ministre de l'intérieur parle d'ensauvagement, tandis que le garde des sceaux dénonce cette rhétorique qui ferait le jeu de l'extrême droite. Le b.a.-ba d'une politique efficace dans tous les domaines, c'est de poser un diagnostic clair et partagé par tous. Nous en sommes très loin ... Même vos ministres les plus importants ne sont pas d'accord entre eux le garde des sceaux recycle la vieille idée socialiste du sentiment d'insécurité, évoquant même un fantasme : il ne doit pas beaucoup sortir des beaux arrondissements de Paris La réalité, monsieur le Premier ministre, c'est que, avec ce jeu de rôle convenu entre justice et intérieur, votre Gouvernement se paie de mots et refuse de regarder la réalité en face, avec courage et bon sens. Vous refusez plus encore d'agir par peur panique de remettre en cause votre idéologie multiculturaliste.

de gendarmerie, on dénombre une agression toutes les deux heures. Au moment de la rentrée scolaire, nous avons rencontré des enfants qui nous ont expliqué que, à l'école, ils n'osent pas dire que leur père est policier, par peur d'être agressés

jusqu'alors écartées. Malgré tout, la situation demeure alarmante : 75 % des agences de voyages pensent déposer le bilan dans les prochains mois et les réservations ont chuté de 50 %, alors que le secteur représente 9 % de notre PIB et 2 millions d'emplois directs et indirects. Au regard de ces enjeux, le plan de soutien à l'activité du secteur présenté en mai dernier, de 18 milliards d'euros, ainsi que les 50 milliards d'euros alloués au tourisme dans le plan France Relance, ne rassurent pas complètement le secteur, inquiet à l'approche de l'annonce de restrictions supplémentaires sur les déplacements et les rassemblements. Les incertitudes qui entourent l'exonération des charges sociales et patronales et la perte de chiffre d'affaires de l'ordre de 73 % subie par les entreprises de transport touristique annoncent une fin d'année très difficile.

locaux. Ainsi, les régions Normandie et Bretagne se sont associées à hauteur de 85 millions d'euros au plan de sauvetage de l'entreprise Brittany Ferries, alors que l'État n'a avancé qu'une aide de 15 millions d'euros. Il est inquiétant de constater que le sauvetage de ce fleuron du pavillon national,

visait à permettre, avant tout, la reprise des trajets domicile-travail. L'offre de transport liée au tourisme a repris cet été, dans le strict respect des gestes barrières, afin d'accueillir de potentiels touristes. le maintien de la fermeture de certaines frontières et les mesures de septaine ou de quatorzaine ont compliqué la reprise du trafic touristique. S'agissant de Brittany Ferries, la décision unilatérale de quatorzaine des autorités britanniques a contraint la majorité des navires à rester à quai.

Voilà près de trente ans que le Haut-Karabakh tente de protéger ses terres ancestrales, alors que l'Azerbaïdjan s'enfonce dans la dictature- rappelons que le régime d'Aliyev est l'un des plus répressifs de la planète Dans ces conditions, on imagine le sort réservé aux Arméniens du Haut-Karabakh, avec la complicité du président Erdogan. Erdogan qui marchande ses migrants, massacre les Kurdes, que nous avons abandonnés, viole les espaces aérien et maritime grecs, qui occupe depuis 1974 Chypre, État de l'Union européenne, tente de déstabiliser encore plus la Libye et la Syrie, souffre d'amnésie dès que l'on parle du génocide des Arméniens et clame sa volonté de reformer l'Empire ottoman, Erdogan dont le régime va jusqu'à envoyer des djihadistes pour tuer des Arméniens On le sait : le président Erdogan cherche, pour masquer ses échecs, à s'offrir comme trophée l'Artsakh, puis l'Arménie, et à poursuivre le génocide culturel et ethnique des Arméniens. Rester neutre face à l'injustice, c'est choisir son camp ! C'est pourquoi la neutralité et l'impartialité ne sont ni acceptables ni responsables : elles reviendraient à soutenir l'agresseur. Lorsque des innocents sont massacrés par des armes interdites, nous ne pouvons rester neutres. Non, la France ne peut pas abandonner son allié, sa soeur : l'Arménie. les Arméniens serait nous renier ; les ignorer, nous trahir. L'indignation est nécessaire, mais ne sauve pas des vies. Il faut agir ! Il est urgent de sanctionner la Turquie et l'Azerbaïdjan, de mettre en place de vraies sanctions économiques, de rappeler nos ambassadeurs à Ankara et à Bakou, cesser tout processus d'adhésion de l'Union européenne avec la Turquie et de lui dire qu'elle n'a plus sa place dans l'OTAN. Il faut encore demander aux forces internationales d'intervenir au sol en Artsakh pour garantir la paix et reconnaître enfin l'État indépendant Artsakh, seul à même de protéger sa population. Un nouveau génocide se met en place, et l'on ne pourra pas dire que l'on ne savait pas. Une partie de l'histoire de l'humanité est en train de s'écrire : faisons en sorte qu'elle ne s'écrive pas sans l'Europe et sans la France

de la Libye au Haut-Karabakh en passant par la Méditerranée orientale, l'Irak et Varosha. Venant d'un État membre de l'Alliance atlantique, c'est particulièrement grave. Nous n'acceptons pas cette logique globale du fait accompli.

par Ankara de mercenaires syriens contribue aussi à l'internationalisation du conflit et fait peser une lourde menace sur la région. Dans cette circonstance, nous devons agir vis-à-vis de la Turquie, en demandant des clarifications

Si nous revenions sur nos engagements de responsables des accords de 1994 et du groupe de Minsk, nous créerions les conditions permettant à la Turquie de remettre en cause l'impartialité

des solidarités et de la santé, à la veille de la journée nationale de mobilisation dans la santé, je veux relayer ici les inquiétudes, le découragement, voire la colère des personnels soignants de l'hôpital public, mais aussi des établissements médico-sociaux. Avec la progression de l'épidémie de covid et l'arrivée de la deuxième vague, vous avez annoncé l'ouverture possible de 12 000 lits de réanimation. Mais vous n'avez pas précisé quels moyens humains supplémentaires seraient prévus pour prendre en charge les malades. Les personnels soignants manqueront, car non seulement ils quittent aujourd'hui l'hôpital public, mais les recrutements sont de plus en plus difficiles. Et ce ne sont pas les mesures du Ségur de la santé qui rendront ces métiers attractifs, ni les annonces de renoncement aux congés qui motiveront les personnels. Je tiens à insister sur la situation particulière des personnels des établissements sociaux et médico-sociaux, exclus des récentes revalorisations salariales. Ce sont près de 40 000 agents de la fonction publique hospitalière qui ne bénéficieront pas du bonus de 183 euros

comment comptez-vous répondre aux attentes de ces personnels, de tous ces hommes et de toutes ces femmes dont le dévouement et le grand professionnalisme ne sont plus à démontrer, mais qui sont aujourd'hui épuisés et inquiets ?

Monsieur le ministre, je ne voudrais pas vous manquer de respect, mais entendez-vous les alertes des professionnels de santé ? Entendez-vous leur inquiétude, au-delà de leur colère ? Oui, leur inquiétude face à la deuxième vague qui arrive,

pas un mois ne passe sans que je sois contacté par des élus désespérés par des installations illicites sur leur commune et hors d'état de lutter contre celles-ci, qui s'accompagnent la plupart du temps de nombreuses incivilités. La situation n'est plus soutenable pour les élus, mais aussi pour les agriculteurs et les chefs d'entreprise qui font face, eux aussi, à ces installations illicites. L'État a bien évidemment des devoirs envers ces communautés, mais ces dernières en ont aussi envers la société : elles doivent notamment participer au vivre-ensemble et ne pas se prévaloir uniquement de leurs droits. En l'absence de respect de ces règles, des mesures et sanctions efficaces et dissuasives doivent être prises. Pour améliorer la gestion de ces situations, ce qui est souhaitable pour tous, et atteindre un certain niveau d'apaisement, plusieurs leviers s'offrent au Gouvernement. J'espère, madame la ministre, que vous saurez les saisir. Tout d'abord, il me paraît important d'organiser une évaluation de l'application de la loi n° 2018-957. Cette démarche permettrait, dans un premier temps, de mieux se rendre compte des faiblesses, mais aussi des forces de ce texte.

à affirmer que ces mesures sont pleinement satisfaisantes. Madame la ministre, quelle sera la position du Gouvernement pour accompagner les élus confrontés à ces situations qui restent intenables ? Très

le maire dispose d'une aire d'accueil conforme au schéma départemental d'accueil des gens du voyage, il peut désormais interdire le stationnement en dehors des terrains aménagés sur sa commune, même si elle appartient à une intercommunalité.

S'agissant de vos propositions, monsieur Pellevat, je rappelle que les préfectures établissent déjà chaque année un bilan des grands passages estivaux des gens du voyage, pour faire état des difficultés qu'elles ont pu rencontrer.

obligatoire leur permet de se confronter à la réalité concrète du travail, mais aussi, pour certains, de préparer déjà leur projet d'orientation. Nous connaissons tous le contexte sanitaire actuel : il est inquiétant. Nous saisissons tous la dimension économique de la crise : elle est catastrophique. de nombreuses entreprises luttent pour leur survie et qu'associations comme collectivités territoriales se concentrent sur les actions de solidarité en faveur des plus démunis, elles n'ont pas le temps de se pencher sur des demandes de stages aussi brefs- même si quelques initiatives locales, comme celles du conseil régional d'Île-de-France et de mon département, promettent d'en satisfaire quelques centaines.

le Gouvernement retire de l'ordre du jour du Sénat le projet de loi prorogeant le régime transitoire institué à la sortie de l'état d'urgence sanitaire. Il demande en conséquence que l'ordre du jour de cet après-midi reprenne pour l'examen du projet de loi relatif à la prorogation des chapitres VI à X du titre II du livre II et de l'article L. 851-3 du code de la sécurité intérieure et du projet de loi organique relatif au Conseil économique social et environnemental, et que l'examen de ce dernier se poursuive ce soir et, éventuellement, demain matin.

La séance est reprise. J'informe le Sénat qu'une candidature pour siéger au sein de la commission spéciale sur le projet de loi relatif à la bioéthique a été publiée. Cette candidature sera ratifiée si la présidence n'a pas reçu d'opposition dans le délai d'une heure prévu par notre règlement. Mes chers collègues, par lettre en date de ce jour, le Gouvernement, à la suite des échanges intervenus en conférence des présidents le 7 octobre dernier, demande l'inscription à l'ordre du jour du jeudi 5 novembre au matin d'une série de questions orales.

devant votre noble assemblée. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la prorogation des chapitres VI à X du titre II du livre II et de l'article L. 851-3 du code de la sécurité intérieure

Il s'agissait alors de sortir de l'état d'urgence, car, chacun en convenait, cet état d'urgence n'avait pas vocation à être permanent. Il s'agissait aussi de maintenir un niveau extrêmement exigeant de sécurité pour les Français, car la menace reste prégnante la lutte contre le terrorisme demeure bien évidemment une priorité nationale. Pour cela, la loi SILT a mis en place des outils nouveaux et adaptés, garantissant un équilibre entre la nécessaire efficacité des actions antiterroristes et la préservation des libertés publiques.

que nos efforts ne doivent pas être relâchés et que nous devons collectivement continuer à agir avec la plus grande détermination contre le terrorisme islamiste.

Je tiens aussi à dire devant la représentation nationale que, depuis 2017, trente-deux attentats ont été déjoués par nos services, c'est-à-dire en moyenne un par mois, dont un encore au tout début de cette année.

interpeller les individus dangereux ou les surveiller, et qui parfois mettent leur vie en péril pour éviter les projets meurtriers. La loi SILT a permis à ces services de continuer à disposer, après la fin de l'état d'urgence, d'un cadre législatif efficace, adapté et validé par le Conseil constitutionnel. L'autorité administrative- préfet ou ministre de l'intérieur, selon les cas -s'est vue reconnaître des compétences nouvelles, strictement proportionnées à l'état de la menace, s'exerçant toujours sous le contrôle du juge et dans le seul objectif de prévenir des actes de terrorisme.

dans lesquels se tiennent ou circulent des idées incitant à la commission ou faisant l'apologie d'actes de terrorisme, et d'édicter à l'encontre d'individus présentant un niveau de menace caractérisée pour la sécurité et l'ordre public des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance, ou Micas. Il s'agit, enfin, de pouvoir solliciter du juge judiciaire l'autorisation de procéder à la visite d'un lieu fréquenté par de tels individus.

dans le même temps, 334 mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance ont été notifiées, dont 60 sont encore actives à ce jour ; 175 visites domiciliaires ont été réalisées. Ces mesures ont toujours été utilisées de manière ciblée et proportionnée, sous le contrôle du juge. Conformément à l'article L. 22-10-1 du code de la sécurité intérieure instauré par l'article 5 de la loi dite SILT, le Parlement a été informé sans délai de la mise en oeuvre de chacune de ces mesures.

Ainsi, depuis 2015, trois traitements automatisés ont été autorisés par M. le Premier ministre, après un avis favorable de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. La délégation parlementaire au renseignement a été rendue destinataire d'un rapport classifié au niveau « confidentiel défense qui décrit la nature de l'apport opérationnel de ces traitements automatisés. Ces derniers ont tout à la fois permis de détecter des contacts entre des individus porteurs d'une menace terroriste, d'obtenir des informations sur la localisation d'individus en lien avec cette menace, de mettre à jour des comportements d'individus connus des services de renseignement et nécessitant des investigations plus approfondies, enfin d'améliorer la connaissance des services sur la manière de procéder des individus de la mouvance terroriste.

Les mesures dont il vous est proposé de prolonger l'application par le présent projet de loi présenté par le Gouvernement constituent donc des outils opérationnels indispensables pour les services spécialisés dans la lutte contre le terrorisme. Ils ont été mis en oeuvre sous le contrôle attentif du juge judiciaire et administratif et, pour certains d'entre eux, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, avis que le Gouvernement a toujours- j'y insiste -suivis. Ils font l'objet d'un échange permanent avec le Parlement, sous la forme d'une information en temps réel et d'une évaluation régulière que le Gouvernement a strictement respectées. Ces dispositifs ont démontré toute leur pertinence dans la prévention de la menace terroriste. C'est également ce que conclut la mission de contrôle mise en place par le Sénat dans son rapport de février dernier, après trois années d'expérimentation. Je relève que la mission sénatoriale estime que la loi a fait l'objet d'une mise en oeuvre équilibrée et conforme à l'esprit du législateur. Elle souligne aussi qu'il existe un consensus de l'ensemble des acteurs, judiciaires comme administratifs, sur l'efficacité et l'utilité des quatre mesures introduites dans la loi SILT dans un contexte de menace extrêmement élevée et à un moment où nous savons que le terrorisme peut frapper partout sur le territoire national. La mission de contrôle, monsieur le rapporteur, s'est en conséquence prononcée en faveur de la pérennisation de ces mesures. Vous-même avez donc logiquement repris les conclusions

Les services de renseignement placés sous mon autorité y étaient prêts. Le ministère de l'intérieur, le ministère des armées et l'ensemble des membres du Gouvernement y étaient prêts. Mais la mobilisation nationale rendue nécessaire par la gestion de la crise sanitaire a fait obstacle à cette discussion parlementaire. Le contexte n'a pas permis aux débats, dans chacune des deux chambres, de se tenir de manière sereine, argumentée et efficace. Or les sujets dont nous parlons sont essentiels pour la sécurité des Français. Ils touchent aux libertés fondamentales. Ils méritent d'être discutés avec la sérénité et le temps nécessaires. Aussi, compte tenu de la sensibilité et de la complexité des dispositions en question, il a semblé opportun au Gouvernement de se donner du temps et de reporter d'un an le débat de fond que nous devions avoir cette année. Pour que ce débat puisse avoir lieu, pour que des dispositions aussi fondamentales ne soient pas entachées de la critique d'un débat démocratique insuffisant, pour qu'elles soient acceptées par l'ensemble de l'opinion, pour que le Conseil constitutionnel puisse les valider, alors qu'elles sont essentielles pour la sécurité du territoire national et pour chacun des Français, j'estime, monsieur le rapporteur, sans vous mettre en difficulté sur le fond, mais en exprimant une légère réserve sur la forme, que la pérennisation ainsi votée serait prématurée.

Les juridictions nationales tireront toutes les conséquences de cette décision européenne. Il nous faudra pouvoir en éclairer le Parlement et examiner avec lui les conséquences potentielles qu'il conviendrait d'en tirer dans la loi. Nous ne sommes donc pas prêts pour les introduire dans le texte que nous présentons aujourd'hui

comme avant, si j'ose dire. Les préfets, les forces de sécurité intérieure et les services de renseignement continueront à se servir des outils qu'ils considèrent, de manière unanime, comme nécessaires à leur action. La mobilisation du Gouvernement pour lutter contre le terrorisme est très forte, et je sais qu'elle est soutenue par la quasi-intégralité des mouvements politiques représentés au Sénat, singulièrement par la majorité sénatoriale qui a, chaque fois, apporté son soutien aux dispositions proposées par le gouvernement d'Édouard Philippe, puis celui de Jean Castex. C'est conscient de la prégnance de la menace terroriste que, depuis 2017, à la demande du Président de la République, le Gouvernement a oeuvré avec une très grande détermination au renforcement des dispositifs pour lutter contre le terrorisme islamiste. Nous l'avons fait en continuant- avec le soutien du Parlement et, en particulier, celui du Sénat -à augmenter les moyens mis à la disposition des services spécialisés en matière de lutte antiterroriste, notamment les services de renseignement.

Ceux de la DGSI ont par exemple doublé entre 2015 et aujourd'hui. La lutte contre le terrorisme exige en effet une mobilisation totale et l'unanimité nationale. Sous l'autorité du Président de la République et du Premier ministre, avec l'engagement de l'ensemble des forces de sécurité et des services de renseignement, avec l'appui du ministère de la justice, nous mènerons un combat sans relâche. Nous ne renoncerons jamais à traquer les ennemis de la République, qui attaquent par la terreur notre identité, notre mode de vie et nos valeurs : la liberté d'expression, la liberté de culte, la liberté de conscience, la laïcité, l'égalité entre les femmes et les hommes.

C'est également pour moi l'occasion de remercier les membres de la commission des lois, quelle que soit leur appartenance politique, mais aussi ceux de la délégation parlementaire au renseignement et de la mission d'information commune sur l'évaluation de la loi relative au renseignement, de la qualité du travail mené en commun depuis plusieurs mois avec mes prédécesseurs Gérard Collomb et Christophe Castaner, et avec moi-même.

depuis maintenant plusieurs années à une menace terroriste élevée, durable, qui s'est malheureusement concrétisée par plusieurs attentats spectaculaires entraînant de très nombreuses victimes blessées, tuées, voire massacrées de manière barbare, comme cela s'est produit au Bataclan. Le dernier exemple en date est l'attaque perpétrée- vous y avez fait allusion, monsieur le ministre -contre les anciens locaux de, à la suite de laquelle deux personnes ont été La menace est multiple, soudaine ou organisée, individuelle ou groupée, bien armée ou non. Grâce à l'efficacité de nos services et aux mesures exceptionnelles qui ont été prises par le Gouvernement, avec l'appui du Parlement, de nombreux attentats ont pu être déjoués. Je veux m'associer, monsieur le ministre, à la gratitude que vous avez exprimée vis-à-vis des services de police, de gendarmerie de police, de gendarmerie et, bien sûr, de la DGSI. Je suis moi-même fils d'un policier qui était spécialisé dans le renseignement : je sais la part d'abnégation et de dévouement qu'il faut pour exercer ce type de métier. Partant de ce constat, ce n'est vraiment pas le moment de baisser la garde. Nous ne pouvons pas nous satisfaire du risque d'une nouvelle attaque terroriste qui plane tous les jours sur la France. Rappelons qu'il n'y a pas si longtemps, en 2018, 30 % des Français estimaient que le terrorisme était le problème le plus important de notre société, classant cette préoccupation en tête de toutes les autres. Aujourd'hui encore, malgré la période exceptionnelle d'épidémie que nous traversons, cette préoccupation reste prégnante dans notre pays. Le Gouvernement et la représentation nationale doivent donc prendre la mesure de la demande et y répondre. Bien évidemment, nous sommes en phase sur cette question.

Ces quatre mesures temporaires- et c'est bien sur l'initiative de la Haute Assemblée qu'elles ont ce caractère -arrivent à échéance le 31 décembre prochain. Cette échéance était connue depuis longtemps.

lesdites mesures, puisque nous étions d'accord sur l'objectif à atteindre. À la même date arrivera à son terme l'expérimentation de la technique dite « de l'algorithme », technique de renseignement qui consiste à imposer la mise en oeuvre sur les réseaux des opérateurs de communications électroniques de programmes informatiques qui analysent les flux de données, en vue de détecter les connexions susceptibles de révéler une menace terroriste ou du prosélytisme. Cette technique ayant suscité beaucoup de craintes lors de son adoption, elle n'a donc, elle aussi, été autorisée par le législateur qu'à titre expérimental. Le débat sur la nécessité de pérenniser ou non ces dispositions aurait dû intervenir dans le courant de l'année 2020. Je vous l'ai dit, nous nous y étions préparés. Pour ma part, j'ai remis deux rapports d'évaluation très explicites Vous l'avez indiqué il y a quelques minutes, le Gouvernement a estimé que la crise sanitaire que nous traversons depuis plusieurs mois risquait de bousculer le calendrier parlementaire et d'empêcher la tenue d'un débat serein au Parlement. Objectivement, nous pensons que ce n'est pas le cas, et c'est là une divergence que nous avons avec vous.

Vous aviez initialement prévu une prorogation d'un an jusqu'au 31 décembre 2021. L'Assemblée nationale, qui a examiné le projet de loi à la fin du mois de juillet, a porté cette durée à sept mois, ce qui supposerait que le Parlement se prononce de nouveau avant l'été 2021, avant le 31 juillet 2021

Je pense pourtant qu'il s'agit d'une nécessité pour maintenir un niveau de vigilance renforcée face à une menace de plus en plus difficile à détecter et nous prémunir face aux risques d'attentats terroristes.

Cette prolongation nous a paru justifiée, moins par le contexte sanitaire et par la conjoncture que par les premiers éléments d'évaluation de l'expérimentation, qui ont été transmis au Parlement à la fin du mois de juin, faisant état de premiers résultats encourageants. Évidemment, sur ce type de sujet très sensible, il faut trouver le bon équilibre pour préserver les libertés. Ainsi, les trois algorithmes déployés par les services de renseignement auraient permis d'identifier des individus qui leur étaient jusqu'alors

la commission des lois n'a en revanche pas suivi la position du Gouvernement et de nos collègues députés. Nous ne nous opposons évidemment pas au maintien des mesures de la loi SILT, mais nous estimons que le report du débat sur leur pérennisation, ainsi que sur les éventuels ajustements à y apporter, n'est pas justifié,

Nous ne voulons évidemment pas porter une atteinte disproportionnée aux droits et aux libertés : ce n'est certainement pas la vocation du Sénat. Le Conseil constitutionnel a d'ores et déjà validé de nombreuses dispositions Notre commission, tout en pérennisant les mesures de la loi SILT, a souhaité proposer quelques évolutions qui sont, somme toute, assez consensuelles pour l'ensemble des acteurs de la lutte contre le terrorisme, afin de les rendre plus efficaces. Elles sont au nombre de trois

élargir les possibilités de saisie informatique dans le cadre d'une visite domiciliaire au cas où l'occupant des lieux ferait obstacle à l'accès aux données présentes sur un support ou un terminal informatique. Monsieur le ministre, ces modifications, qui ont d'ailleurs fait l'objet d'un large consensus avec vos services, sont essentielles et répondent à des besoins exprimés clairement pour une meilleure efficacité. Nous pensons donc qu'il ne faut pas reporter leur mise en oeuvre et assumer dans les plus brefs délais. Avant de clore mon propos, je tiens à vous faire part de notre inquiétude persistante. Vous le savez, nous avons mené plusieurs missions sur la gestion des condamnés terroristes sortant de détention. Même s'il ne s'agit pas de l'objet du présent projet de loi, raison pour laquelle je n'ai pas déposé d'amendement à ce sujet,

Le Sénat a toujours fait preuve de responsabilité dans le strict respect des libertés individuelles : c'est cet esprit qui doit nous conduire à approuver le texte tel que la commission des lois

qui proroge l'article L. 851-3 du code de la sécurité intérieure relatif à la technique de renseignement dite « de l'algorithme ». À travers mon intervention, je défends aussi la position de la délégation parlementaire au renseignement, la DPR, que j'ai eu l'honneur de présider l'an passé. Nous sommes plusieurs dans cette enceinte à nous souvenir des débats nourris que nous avions eus, ici même, en 2015 lors de l'adoption de ce dispositif expérimental. Certains collègues souhaitent rouvrir ce débat aujourd'hui. Tel n'est pourtant pas le calendrier prévu. Certes, dans une démocratie, il faut toujours garder le cap d'un équilibre entre l'efficacité de la lutte contre le terrorisme et la préservation des libertés publiques, mais, en l'espèce, le projet de loi que nous examinons ce jour ne pose aucune question nouvelle en matière de libertés publiques, comme l'a très bien exposé le rapporteur au fond, Marc-Philippe Daubresse. Je voudrais brièvement rappeler les limites que le législateur a fixées en 2015 à cette technique, et les garanties qui en découlent. Citons les principales. Premièrement, l'utilisation des algorithmes doit avoir un objet très ciblé, puisqu'il ne s'agit que de la lutte contre le terrorisme. un dispositif tout entier soumis au contrôle de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, la fameuse CNCTR, doit être mis en oeuvre. Je rappelle l'importance

Troisièmement, l'algorithme ne traite que des données de connexion, et non les données de contenu. Du reste, nous avons abordé ce point dans le rapport de la DPR que je viens de remettre au Président de la République. Quatrièmement, ce dispositif produit des résultats anonymisés.

Naturellement, on peut comprendre que la nouveauté du dispositif ait suscité des craintes en 2015. On voit que la réalité est en fait beaucoup plus modeste. À vrai dire, l'enjeu opérationnel des trois algorithmes qui existent aujourd'hui est précisément de restreindre les résultats aux seuls éléments pertinents et utilisables. On est donc loin du contrôle de masse indiscriminé évoqué à l'époque. Il me semble, enfin, que, lorsque nous légiférons sur ces questions, il nous faut garder à l'esprit le caractère encore récent de cette technique.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

Nous sommes en effet d'accord sur le contenu des quatre prérogatives spécifiques, qui ont été instaurées en 2017 à l'issue de l'état d'urgence, c'est-à-dire les visites domiciliaires, les mesures individuelles de contrôle administratif, les périmètres de protection et les fermetures de lieux de culte. Le projet de loi prévoit aussi la prorogation de l'utilisation, dans les conditions limitées que vient de décrire le président Christian Cambon, des algorithmes de tri de données permettant le repérage des menées terroristes.

la préparation de ces mesures, disons, de « confortement » des algorithmes est rendue plus difficile par les récentes décisions de justice, qui confirment d'ailleurs une jurisprudence antérieure de la Cour de justice de l'Union pour des motifs qui tiennent beaucoup plus à la protection du consommateur de services informatiques qu'à des préoccupations de sécurité publique et de nature régalienne, affirme que l'on ne peut pas imposer aux opérateurs eux-mêmes de conserver des données pour une durée indéterminée sur instruction des autorités de sécurité publique. Le Conseil d'État aura

de prévoir des mesures de sûreté, certes plus restreintes et plus limitées dans le temps, mais qui permettraient d'encadrer les mouvements des personnes sortant de détention après avoir été condamnées pour terrorisme.

la position de la commission est proche. J'ai eu le privilège de participer à toutes les discussions en matière de législation antiterroriste depuis 2015 : il y a toujours eu un accord entre le Gouvernement,

Nous comprenons la nécessité absolue de sécuriser juridiquement des mesures qui pourraient intervenir au-delà du 31 décembre 2020. Pour autant, nous tenons à préciser que, dans notre esprit, cette prorogation ne vaut pas blanc-seing. Le Parlement doit pleinement exercer sa mission constitutionnelle de contrôle du Gouvernement, dans un domaine où le respect des droits et des libertés est mis en balance avec l'impératif de protection de nos concitoyens. Ainsi, comme l'indiquait à juste titre le Défenseur des droits en 2017 dans son avis sur le projet de loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, l'enjeu est de taille. Il s'agit bien de maintenir « l'équilibre qui fonde le droit pénal entre exigences de sécurité et protection des droits et libertés, et, d'autre part, l'équilibre entre rôle de l'autorité administrative et celui de l'autorité judiciaire. Si nous entendons l'argument de la crise sanitaire qui contraint le calendrier parlementaire, les conditions d'exercice de nos libertés fondamentales valent bien, à notre sens, un débat approfondi. Nous en avons encore eu la preuve hier lorsque nous avons discuté des mesures de sortie de l'état d'urgence sanitaire. Nous ne pensons pas que la succession de textes d'exception doive devenir une habitude. Au contraire, il faut, je le crois, viser une certaine stabilité de notre législation en matière de sécurité intérieure et de renseignement, sans rien céder pour autant à l'angélisme et aux bons sentiments. La commission des lois, suivant son rapporteur, a pérennisé des dispositions d'exception, comme la possible fermeture administrative de lieux de culte. Elle a aussi élargi les conditions de saisie informatique à domicile en cas de refus d'accès aux données, tout en renforçant l'information des autorités judiciaires sur les mesures individuelles de contrôle. Là encore, nous aurons bien sûr besoin d'évaluations ultérieures pour mesurer pleinement l'efficacité et les effets de ces dispositions, dont nous comprenons qu'elles sont indispensables à nos services de police et de renseignement. Mon groupe émet cependant quelques réserves sur l'expérimentation en cours de la technique des algorithmes et sur sa prorogation. Nous prenons bien entendu acte de l'avis favorable de nos collègues de la commission des affaires étrangères. Rappelons toutefois que ces techniques de surveillance, qui font appel à l'utilisation de l'intelligence artificielle, évoluent depuis cinq ans dans un environnement très mouvant sur le plan technologique et dans lequel, de surcroît, notre souveraineté a du mal à se faire valoir. Trois algorithmes différents sont actuellement en vigueur. Le champ d'expérimentation n'est pas le même qu'il y a trois ans et ne sera pas le même dans six mois. En conclusion, En conclusion, nous plaidons pour un renforcement du contrôle parlementaire. La commission des lois pourrait sans doute se saisir utilement d'une réflexion prospective, et ce dans la perspective de l'examen du projet de loi relatif au renseignement de 2021. chers collègues, par raison- à savoir notre attachement à l'ordre républicain et à la sécurité de nos concitoyens -plus que par conviction, le groupe RDSE soutiendra et votera ce texte.

instauraient, une échéance fixée au 31 décembre prochain. Prenant prétexte de la crise sanitaire et considérant, de ce fait, que le Parlement ne disposait pas du temps nécessaire pour débattre des conditions dans lesquelles ces dispositifs doivent être abandonnés, pérennisés ou aménagés, le Gouvernement a souhaité les proroger d'un an.

comme l'indique dans l'une de ses motions le Conseil national des barreaux, « les dispositifs mis en place par la loi dite " SILT ", très intrusifs, qui s'apparentent à des assignations à résidence et des perquisitions contrôlées par l'administration, contournent la procédure judiciaire et les droits de la défense ». Et d'ajouter : « ces dispositifs ont des conséquences très lourdes pour les personnes visées ». En effet, la loi SILT a transformé les assignations à résidence en « mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance » et les perquisitions en « visites et saisies ». Mais il s'agit bien des mêmes mesures liberticides que celles de l'état d'urgence, contournant la justice pénale ordinaire et les protections qui lui sont associées, mesures, dans leur très grande majorité, fondées sur des informations confidentielles, difficiles à contester et qui ouvrent donc la voie à des discriminations. L'état d'urgence n'a malheureusement pas prouvé son utilité pour prévenir les actes de terrorisme et il a été la source de dérives inacceptables, comme les assignations à résidence détournées de leurs objectifs initiaux en étant, par exemple, utilisées à l'encontre de militants écologistes.

En quoi votre rapport nous prouve-t-il que ce régime dérogatoire est nécessaire pour notre sécurité ? Le droit pénal et nos services de renseignement, dont les moyens humains doivent être renforcés, sont largement suffisants Amnesty International a d'ailleurs déjà démontré que les dispositions de la loi pouvaient mener à des violations du droit au respect à la vie privée et familiale, du droit au travail, de la liberté d'aller et venir et du droit à une procédure équitable, en plus des graves conséquences psychologiques En outre, en 2018, lors de l'examen périodique universel de la France à l'Assemblée générale des Nations unies, plusieurs États se sont inquiétés du manque de respect des droits humains dans le cadre de la lutte contre le terrorisme dans notre pays et ont insisté sur la nécessité de mettre en place un mécanisme indépendant de suivi. Quant à l'article 2 du projet de loi, il vise à proroger la disposition expérimentale issue de la loi du 24 juillet 2015 relative au renseignement : la technique de recueil de renseignements algorithmique. Plus que critiquable sur le fond, cette technique apparaît de surcroît inutile, puisque l'analyse en continu des données par les boîtes noires n'aurait permis de détecter qu'une petite dizaine de profils faiblement à risque. La disproportion entre ces résultats et les moyens mis en oeuvre pour écouter et observer la société tout entière est, pardonnez-moi, aberrante ! De plus, dans son arrêt du 21 décembre 2016, la Cour de justice de l'Union européenne a estimé qu'une réglementation nationale prévoyant, à des fins de lutte contre la criminalité, une telle conservation des données constituait en soi une atteinte disproportionnée aux droits fondamentaux. Au moment des débats sur la loi SILT, nous dénoncions déjà la banalisation des mesures d'urgence et la fragilisation de l'État de droit et des libertés fondamentales. Aucune évaluation des dispositifs prorogés n'a été faite. En dépit des décisions de censure de certaines dispositions par le Conseil constitutionnel, ni la nécessité, ni la proportionnalité, ni l'efficacité de telles mesures n'ont été démontrées. Nous restons aujourd'hui convaincus que les vraies réponses à apporter pour lutter contre le terrorisme résident dans les moyens donnés à la justice et aux services de renseignement, plutôt que dans la surenchère en matière législative. Tous les fonctionnaires de terrain en témoignent : les lois ne manquent pas, les moyens oui ! Pour toutes ces raisons, vous l'aurez compris, nous voterons définitivement contre ce projet de loi.

monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues,

et 20 morts depuis 2017, tout en mettant en balance les 32 attaques qui auraient été déjouées. Nous comprenons donc bien les difficultés et le niveau du péril.

aux mesures très précises, et qui ont été ajustées, figurant dans les propositions de la mission de contrôle, notamment l'extension de la fermeture aux lieux connexes

fond conduisent mon groupe à privilégier la pérennisation à la prorogation sèche. Premièrement, notre préférence pour le recours au droit commun. Nous sommes en général très réticents à des mesures d'exception.

mais antérieur à la décision de la Cour de justice de l'Union européenne. Il s'agit d'un document extrêmement technique, expliquant comment ont été sélectionnés les trois algorithmes et exprimant un certain nombre de demandes, notamment sur les données IP et URL. Il est clair

que le texte soit critiquable. C'est la raison pour laquelle j'ai indiqué, en préambule, que mon groupe était à l'aise sur ces sujets. S'il restait pour le ministère de l'intérieur, ou pour le Gouvernement au sens large,

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le

Mais nous fûmes, toutes et tous, stupéfaits par cette violence et par cette haine. Au sein du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, nous sommes fiers de l'action que menèrent, alors, François Hollande et Bernard Cazeneuve. Jamais ils n'ont dévié d'une ligne de fermeté républicaine dans le cadre de l'État de droit. Car la victoire du terrorisme, mes chers collègues, serait que nous changions, que nous ne chérissions plus notre liberté par peur pour notre sécurité, que nous renoncions à « être Charlie », que nous renoncions à être nous-mêmes. Au nom de mon groupe, je souhaite d'abord rendre hommage à celles et ceux qui se sont engagés et qui s'engagent dans cette lutte contre le terrorisme, dans les services de police et de renseignement,

En 2015, avec la loi relative au renseignement et la création de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, nous avons encadré les actions des services de renseignement, en leur donnant des moyens et en adoptant la possibilité de faire des expérimentations par algorithme des données de connexion. En 2016, enfin, une proposition d'introduction de l'état d'urgence dans la Constitution aurait pu permettre

de culte et des périmètres de protection. Compte tenu de la nature de ces mesures administratives, c'est le Sénat, sur l'initiative du président de la commission des lois de l'époque, Philippe Bas, qui a émis le souhait d'une application expérimentale pour trois ans, et le Conseil constitutionnel s'est prononcé dans ce cadre de mesures strictement contrôlées par le Parlement et provisoires.

ou de conservation des données entre la voix et l'image, vous n'en voulez pas dans la deuxième partie. C'est un peu paradoxal

de renforcer les exigences relatives aux motivations de mise en oeuvre d'une visite domiciliaire. Enfin, nous refuserons la suppression des mesures permettant un contrôle parlementaire effectif. de la deuxième partie du texte, nous proposerons d'autoriser la CNCTR à accéder aux fichiers de souveraineté dans le cadre de sa mission de contrôle et de simplifier des dispositions relatives à la conservation des données et aux décisions de la CNCTR,

porter atteinte aux libertés, si nous avions toutes les garanties d'une mise en oeuvre correcte et d'un contrôle parlementaire très pointilleux. Mais il est probable, malheureusement, que nos propositions ne soient pas retenues ... Ainsi, sauf bonne surprise- c'est toujours possible dans un débat parlementaire -, il est également probable que mon groupe soit contraint de voter contre ce texte, à l'issue de nos débats. Mais ... espérons une bonne nouvelle

le niveau de la menace à laquelle la France a été confrontée, en particulier depuis 2015, n'a malheureusement pas faibli. Oui, le risque terroriste est toujours là ! Oui, le danger islamiste est toujours présent ! Le terrorisme islamiste est susceptible de frapper n'importe quand et n'importe où sur notre sol. Le virus n'a pas amoindri la menace, laquelle demeure élevée. La plus grande vigilance reste donc de mise. Bien au contraire, nous constatons les avancées des islamistes dans nos quartiers, des attentats terroristes à bas bruit. On n'en parle presque plus, mais ils rappellent que la menace reste présente partout. En témoigne l'acte de l'assaillant terroriste devant les anciens locaux de, voilà quelques jours. Cette attaque était la quatrième perpétrée sur le sol français depuis le début de l'année. Cette menace va se renforcer encore avec des sorties de prison inquiétantes d'ici à la fin de l'année, 45 détenus condamnés pour terrorisme seront libérés. Au total, on compte encore 5 050 individus condamnés pour terrorisme dans les geôles françaises. Plusieurs dispositions du code de la sécurité intérieure introduites au cours des dernières années pour renforcer l'arsenal de lutte contre le terrorisme ont reçu, compte tenu de leur sensibilité au regard des libertés publiques et individuelles, un caractère temporaire et arriveront à échéance, sauf intervention du législateur, le 31 décembre prochain. Sont tout d'abord concernées quatre dispositions de la loi du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, à savoir les périmètres de protection, la fermeture des lieux de culte, les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance, les visites domiciliaires et saisies, telles que les perquisitions administratives. Est également visée la technique de l'algorithme, consistant à imposer la mise en oeuvre sur les équipements d'opérateurs de communications électroniques et de fournisseurs de services d'accès à internet de programmes informatiques analysant les flux de données, en vue de détecter des connexions susceptibles de révéler une menace terroriste. Au regard des craintes qu'elle a suscitées à l'occasion de l'examen du projet de loi relatif au renseignement au Parlement, cette technique a été strictement encadrée par le législateur et n'a été autorisée qu'à titre expérimental. Initialement fixée au 31 décembre 2018, l'échéance de cette expérimentation a été repoussée de deux ans, en raison des difficultés techniques rencontrées par les services de renseignement pour définir l'architecture et le paramétrage du dispositif. Sauf prorogation ou pérennisation par le législateur, cette mesure prendra donc fin le 31 décembre prochain. La menace terroriste étant toujours prégnante, l'État a besoin de ces outils pour assurer la sécurité des Français. L'objet de ce projet de loi, composé de trois articles, est simple : prolonger d'une année la durée de validité de ces différentes dispositions expérimentales, qui prennent fin simultanément le 31 décembre Les articles 1 et 2 procèdent, respectivement, à la prorogation des dispositions de la loi SILT et de l'article L. 851-3 du code de la sécurité intérieure relatif à l'algorithme. L'article 3, quant à lui, vise à rendre cette prorogation applicable dans certaines collectivités d'outre-mer. Initialement fixée à un an, la durée de ces prorogations a été ramenée à sept mois par l'Assemblée nationale, afin de ne pas retarder excessivement la tenue d'un débat de fond sur les mesures concernées. Je me réjouis que la commission des lois du Sénat ait souhaité pérenniser, sous réserve de certains ajustements destinés à en renforcer l'opérationnalité, plutôt que prolonger les dispositions de la loi SILT, déjà évaluées et à l'efficacité prouvée. Je me félicite également que la commission ait accepté la prorogation simple de l'article L. 851-3 du code de la sécurité intérieure, proposée par le Gouvernement, jugeant qu'il était préférable de reporter le débat sur l'algorithme à une discussion plus large sur la loi relative au renseignement. Avant de conclure, je souhaite rendre hommage aux services de renseignement- cela a déjà été fait -, aux policiers, aux gendarmes, qui font chaque jour un travail exceptionnel pour identifier les menaces, suivre les individus dangereux et faire échouer leurs projets meurtriers.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la tâche qui est aujourd'hui la nôtre est loin d'être aisée, puisqu'il nous est demandé de trouver un précaire équilibre entre la liberté et la sécurité Malheureusement, derrière l'objectif affiché de donner à ceux-ci un cadre de vie serein et apaisé, à l'abri de toute menace terroriste, ce projet de loi ne parvient pas suffisamment à concilier ces deux enjeux essentiels à l'existence d'une société libre et éclairée. En 2017, la loi SILT avait incorporé dans le droit commun des mesures de l'état d'urgence. Pour la première fois, des dispositions d'exception avaient revêtu un caractère général, banalisant au sein de notre législation des mesures de police administrative qui sont loin d'être anodines. Le législateur d'alors ne s'y était pas trompé. Il avait donné à ces mesures un caractère temporaire et avait souhaité limiter leur durée d'application au 31 décembre 2020. Cette échéance arrivant à son terme, l'exécutif s'est tout naturellement saisi de cette question. Mais, alors qu'un débat sérieux aurait dû être mené sur l'abrogation ou la pérennisation de ces mesures, le Gouvernement a préféré prolonger l'expérimentation conduite depuis 2017, estimant que la crise sanitaire pourrait être de nature à biaiser les discussions parlementaires. Ainsi était-il proposé, à l'article 1, de proroger de sept mois des dispositions de la loi SILT conférant à la police administrative des pouvoirs trop importants : pouvoirs, notamment, de définir des périmètres de protection, de déclarer la fermeture temporaire de lieux de culte, d'ordonner des mesures individuelles de contrôle et de surveillance,

pour les algorithmes votés en 2015 et prolongés en 2017. Ceux-ci permettent notamment de détecter les menaces terroristes les réseaux internet et de téléphonie mobile. Il est à déplorer que les travaux conduits en commission des lois n'aient pas été de nature à améliorer ce texte, M. le rapporteur ayant jugé utile de faire voter un amendement qui vise à pérenniser les mesures prévues à l'article 1. Il va sans dire que nous ne pouvons pas considérer positivement cette modification, tant elle fait la part belle au soupçon, à l'arbitraire, aux dérives, à la stigmatisation par l'administration, au détriment

un danger immédiat ou sérieux pour la sécurité nationale. Sans une amélioration drastique de ces dispositifs numériques que vous qualifiez vous-même, monsieur le rapporteur, de « trop peu sophistiqués », et à défaut de résultats plus probants, il n'est pour l'heure pas pertinent de continuer à investir dans ces moyens d'espionnage informatique, ne serait-ce que temporairement, jusqu'au 31 juillet 2021. Monsieur le ministre, mes chers collègues, personne dans cette enceinte ne nie la menace terroriste qui plane et pèse sur notre nation. Il est évident que nous devons doter massivement nos services de renseignement de moyens humains, techniques et financiers. En ce sens, tout doit être fait pour préserver la sécurité de nos concitoyens, mais non à tout prix. Je crains, hélas, qu'en l'état l'exécutif ne fasse fausse route. Sans débat démocratique réel, sans bilans sérieux de ces mesures, celles-ci ne sauraient être prorogées ni pérennisées. Pour ces raisons, le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires votera contre ce texte. La parole

comme le rappelait le garde des sceaux, ministre de la justice, au mois de juillet dernier, à l'occasion de nos débats sur la proposition de loi instaurant des mesures de sûreté à l'encontre des auteurs d'infractions terroristes à l'issue de leur peine, dont j'étais rapporteure, les chiffres sont connus et ils sont inquiétants 260 personnes sont actuellement détenues après une condamnation pour une infraction terroriste en lien avec la mouvance islamiste. Outre ces détenus condamnés, 252 personnes sont en détention provisoire après mise en examen pour des faits de terrorisme. Elles seront jugées dans les mois ou années à venir : 49 procès devraient se dérouler d'ici à 2021. Parmi les condamnés- n'oublions pas ces chiffres

comme le suggère le Gouvernement, en se bornant à proroger des dispositions dont notre mission sénatoriale de contrôle et de suivi de la mise en oeuvre de la loi SILT a dit toute la pertinence et l'efficacité en février dernier Pourquoi attendre un nouveau projet de loi, alors que le texte que nous examinons aujourd'hui tient déjà compte des « évolutions induites par les besoins opérationnels », pour reprendre les termes employés en conseil des ministres le 17 juin 2020 ? Notre rapporteur l'a préconisé, et nous l'avons suivi en commission : les quatre dispositions de la loi SILT doivent être pérennisées, et non seulement prolongées ! Bien sûr, il existe un point d'équilibre entre sécurité et liberté, vers lequel nous devons tendre en permanence. Mais ne détournons pas le regard : notre obligation première est celle d'assurer la sécurité des Français. Si nous ne nous donnons pas les moyens de protéger nos concitoyens, nous aurons en effet beau jeu de leur dire que nous faisons tout notre possible pour garantir leur liberté. L'une des dernières études du Centre d'analyse du terrorisme communiquée au Sénat atteste une fois de plus la gravité de cette question. Elle révèle en effet que le taux de récidive des djihadistes se situe, selon les situations, au-delà de 50 il est souvent probable qu'un islamiste engagé dans une action violente se maintienne dans cette mouvance et récidive. Mes chers collègues, nous avons pris du retard. La lourde censure par le Conseil constitutionnel de la loi instaurant des mesures de sûreté à l'encontre des auteurs d'infractions terroristes que nous déplorons- nous avions pourtant apporté à ce texte un certain nombre de garanties -, nous oblige aujourd'hui à faire preuve de pragmatisme. « Pragmatisme » : j'emploie ce mot à juste titre. Sur d'autres travées, certains nous reprochent parfois de poursuivre une quête illusoire de sécurité absolue, au détriment d'autres libertés. Il n'en est rien. En effet, mes chers collègues, sans sécurité, l'exercice de nos libertés fondamentales est-il possible ? Aussi est-il urgent que nous dotions notre arsenal législatif de suivi des auteurs d'actes terroristes de toutes les mesures qui ont d'ores et déjà démontré leur caractère opérationnel. Pour conclure, je tiens à remercier notre rapporteur, cher Marc-Philippe Daubresse, de la qualité de son travail. Pour l'ensemble des raisons que j'ai évoquées, le groupe Les Républicains votera ce projet de loi tel qu'amendé par la commission des lois.

pour présenter l'amendement n° 3 rectifié. Par la loi SILT de 2017, le législateur a introduit dans le droit commun des mesures administratives liées à l'état d'urgence. Parmi elles, quatre relevaient d'un régime temporaire : la définition des périmètres de protection, la fermeture des lieux de culte, les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance et les visites domiciliaires. Ces mesures arrivant à échéance le 31 décembre 2020, un débat parlementaire aurait normalement dû se tenir, afin d'évaluer leur pertinence et leur proportionnalité. Faisant fi des principes démocratiques de base et du devoir d'information du Parlement, le Gouvernement a décidé de proroger ces dispositions sans véritable évaluation de fond. La droite La droite sénatoriale est allée encore plus loin, puisqu'elle a décidé, en commission, de pérenniser ces mesures, les incorporant définitivement dans le droit commun. Mes chers collègues, nous ne pouvons nous satisfaire d'une telle décision. Les dispositifs introduits dans notre droit par la loi SILT donnent à l'administration des pouvoirs exorbitants, qui bafouent les droits de la défense et contournent le contrôle du juge judiciaire. La sécurité de nos concitoyens est primordiale, mais la lutte contre le terrorisme ne saurait être assurée par le biais de procédés administratifs arbitraires et attentatoires aux libertés publiques individuelles. Ainsi est-il demandé, le présent amendement, que soit supprimé l'article 1 du présent projet de loi. La parole

la pérennisation de ces mesures exceptionnelles qui ont été votées pour trois ans, cette échéance ayant été adoptée sur l'initiative de notre assemblée.

un vrai consensus se dessine, du côté aussi bien de l'autorité administrative que de l'autorité judiciaire, pour que ces mesures puissent perdurer. Enfin- je l'ai dit -, le Conseil constitutionnel a confirmé la conformité à la Constitution de ces mesures. Il n'y a par conséquent pas lieu de s'inquiéter

vise à sécuriser le cadre légal des périmètres de protection en tendant à inscrire dans la loi, par souci de lisibilité, la réserve d'interprétation que le Conseil constitutionnel avait émise concernant les opérations qui sont menées

demander qu'un décret en Conseil d'État établisse un référentiel des pièces types permettant de motiver les requêtes des visites domiciliaires et saisies et d'étayer les critères prévus au présent article. C'est une demande des juges

à l'amendement n° 7, nous sommes d'accord sur le fond, mais pas sur le vecteur. M. Leconte propose un décret en Conseil d'État. Je recommandais, dans mon rapport, la mise en place d'un référentiel pour améliorer la motivation des requêtes des visites domiciliaires.

Cette technique de renseignement, que nous dénonçons depuis 2015, n'a formellement fait l'objet que d'une application relativement faible et limitée : à la fin de l'année 2019, trois algorithmes auraient été mis en oeuvre depuis leur légalisation. Selon un rapport confidentiel, les techniques en question n'auraient même jamais permis d'empêcher un seul acte terroriste. Pouvez-vous infirmer ou confirmer cette information, monsieur le ministre ? L'analyse en continu des données par les boîtes noires n'aurait jamais permis de détecter qu'une petite dizaine de profils faiblement à risque. Là encore, monsieur le ministre, pouvez-vous infirmer ou confirmer cette information ?

En outre, dans un arrêt du mois de décembre 2016, la Cour de justice de l'Union européenne a estimé qu'une réglementation nationale prévoyant, à des fins de lutte contre la criminalité, une telle conservation des données constituait en soi une atteinte disproportionnée aux droits fondamentaux. Cette jurisprudence, qui sera sans doute prochainement confirmée par l'issue donnée aux renvois préjudiciels effectués notamment par le Conseil d'État français, est selon nous l'énième signal du caractère dangereux de cette technique de renseignement intrusive et inefficace qui n'aurait jamais dû être légalisée, même sous

discussion générale. Il s'agit de dispositifs expérimentaux, et le Gouvernement lui-même propose de prendre le temps de bien réfléchir, de poursuivre l'expérimentation et d'avoir une discussion approfondie sur la loi Renseignement.

connexion par algorithme. Toutefois, depuis, j'ai pu constater à quel point en particulier la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement était impliquée dans sa mission de contrôle, qu'il s'agisse des avis qu'elle devait rendre sur les demandes pour mettre en place une technique de renseignement ciblée

Mais nous défendrons ultérieurement un certain nombre d'amendements visant à améliorer le fonctionnement de cette Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement pour qu'elle remplisse au mieux sa mission et puisse nous donner toute confiance sur la manière dont les services de renseignement utilisent les moyens qui sont à leur disposition.

du code de la sécurité intérieure, la durée maximale de conservation des données collectées par les dispositifs de captation de paroles avant destruction est de trente jours à compter de leur recueil pour les paroles prononcées à titre privé et celle des données de captation d'images

et rend difficile le travail à la fois des services de renseignement, mais aussi de la CNCTR. Par souci de simplification et de cohérence du cadre légal en vigueur, le présent amendement tend à instaurer une durée maximale de conservation unique pour ces deux catégories de données qui sont souvent récupérées en même temps. Quel

aux fichiers de souveraineté. Cet accès s'applique notamment aux traitements intéressant la sûreté de l'État dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, y compris lorsque ces traitements comportent des éléments communiqués par des services étrangers

pour avoir un débat de fond dans le cadre de la loi Renseignement. Avis défavorable.

ainsi que de la loi organique n° 2010-837 et de la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 prises pour son application, la commission des affaires économiques a émis, lors de sa réunion de ce jour, un avis favorable- 33 voix pour -à la nomination de M. Philippe Mauguin à la présidence de l'Institut national de la recherche, de l'agriculture et de l'environnement.